le décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire, à compter du 1 juillet 2020, a été porté à la connaissance du Sénat. En conséquence, je constate que la session extraordinaire est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation ? ... Le

mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris la disparition, le 25 juin, de notre ancien collègue Patrice Gélard, qui fut sénateur d'un département cher à votre coeur, monsieur le Premier ministre, la Seine-Maritime, de 1995 à 2014. Diplômé de « Langues O' », docteur en sciences politiques et en études slaves, agrégé de droit public, Patrice Gélard fut d'abord un professeur de droit constitutionnel passionné qui a marqué des générations d'étudiants. Universitaire de renom, il fut doyen de la faculté de droit de l'université de Rouen, puis doyen de la faculté des affaires internationales de l'université du Havre. Engagé en politique au Rassemblement pour la République (RPR), il fut aussi un élu local profondément ancré dans son département. Il fut conseiller municipal du Havre de 1983 à 2008, conseiller général de 1994 à 2001, adjoint au maire du Havre de 2001 à 2008, vice-président de la communauté d'agglomération du Havre de 2001 à 2014, maire de Sainte-Adresse 2008 à 2014, dont peu savent qu'elle fut la capitale de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, symbole de résistance. Élu sénateur en 1995, puis réélu en 2004, Patrice Gélard s'investit fortement dans sa mission de législateur et devint rapidement un pilier de la commission des lois, dont il fut vice-président à Constitutionnaliste éminent, il fut le rapporteur infatigable de plusieurs projets de loi constitutionnelle, de multiples projets de loi concernant nos institutions et de diverses réformes de notre règlement, mais aussi de grands textes de droit civil.

Grand spécialiste des institutions de l'Union soviétique et des pays de l'Est, il fut longtemps le président du groupe d'amitié France-Russie, distingué dans l'ordre de l'Amitié russe France et la Russie. Patrice Gélard a fait bénéficier nos débats de son exceptionnelle érudition, de sa grande rigueur intellectuelle, de son indéfectible liberté d'esprit et de son remarquable talent d'orateur, dans toutes les langues.

qui se consacrait à d'autres passions moins connues : l'écriture, le dessin, la peinture, le théâtre et la collection de soldats de plomb ... Je souhaite exprimer notre sympathie attristée et notre profonde compassion à son épouse Marie-Claude, à ses enfants Sophie, fonctionnaire du Sénat,

le décès de Patrice Gélard. Il était un sénateur respecté et estimé dans cette assemblée ; il était, pour ses amis havrais, un exemple de culture, un exemple d'engagement local à la fois tranquille et résolu

d'aucun autre homme ou femme politique. Jamais ! Et c'est assez rare ! Il était malicieux, il était fidèle. Je pense à son épouse, à ses enfants, bien sûr, et je pense aussi à son ami Antoine Rufenacht.

Et puis il était un universitaire, un universitaire non pas égaré dans le monde politique, mais qui pensait que le savoir et la connaissance devaient être aussi l'un des fondements de l'action politique. Monsieur le président, je partage très vivement l'émotion que vous avez exprimée, et je sais que, samedi, à Sainte-Adresse, dans l'église Saint-Denis, nous serons nombreux à lui dire à la fois notre amitié, notre estime et notre admiration.

L'énergie nucléaire, dont cette centrale est emblématique, a permis aux Français de bénéficier d'une électricité deux fois moins chère qu'en Allemagne. Elle a permis à la France de n'émettre que 1 % des émissions mondiales de CO2, la plaçant très loin devant son voisin allemand. Elle a, enfin, fortement bénéficié à l'emploi et à l'attractivité de la région alsacienne. La décision de M. Hollande que vous mettez en oeuvre aujourd'hui, ce sont près de 2 000 emplois locaux qui vont disparaître, sans aucune concrétisation du plan de reconversion promis par l'État ; ce sont 400 millions d'euros d'indemnités que l'État devra verser à EDF, comme l'a cruellement rappelé la Cour des comptes dans un rapport particulièrement sévère ; ce sont entre 6 et 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an, le repli vers l'éolien et le solaire ne pouvant conduire qu'à importer davantage d'énergie carbonée

Madame la ministre, la décision que vous avez prise aura des conséquences particulièrement négatives. Cette décision n'est pas économique : la facture énergétique des Français et des entreprises françaises va largement progresser. Elle n'est pas sociale : vous pénalisez très fortement tout un bassin d'emploi. Elle n'est évidemment pas écologique : vous privez notre pays d'une énergie décarbonée, et c'est visiblement un avis partagé par M. le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Madame la ministre, pouvez-vous donc nous dire ce qui a vraiment motivé ce choix ?

Avec cette décision, nous tenons nos promesses. Nous transformons en profondeur notre modèle énergétique et nous accompagnons les Français et les territoires dans cette transformation. Avec l'arrêt des deux réacteurs de Fessenheim, nous engageons la réduction à 50 % de la part du nucléaire d'ici à 2035 tout en développant massivement les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'un système électrique plus diversifié est un système plus plus résilient. C'est pour cela que nous allons multiplier par deux la part de l'éolien et par cinq la part du photovoltaïque dans les dix ans. Mais, dans le même temps, le Gouvernement est particulièrement vigilant à l'accompagnement des salariés et des territoires. S'agissant des salariés d'EDF, ils seront tous reclassés au sein du groupe. Ils sont sauvés ! S'agissant des salariés des sous-traitants, une cellule de reclassement est en place pour les accompagner. Concernant la reconversion du territoire, 35 millions d'euros ont déjà été engagés, même s'il est vrai que la crise a conduit à prendre du retard dans la la mise en place des différents dispositifs. Je voudrais souligner l'annonce récente d'un projet d'implantation d'une usine de biocombustibles, qui pourrait créer 700 emplois dans le territoire. donc assurée, madame la sénatrice, que notre politique énergétique s'inscrit pleinement dans le respect de l'accord de Paris et que nous accompagnons les Français et les territoires dans la transition.

qui puisse être à la hauteur du défi que représente l'arrêt des réacteurs nucléaires. À cet égard, je regrette que le Gouvernement ait refusé la feuille de route que le Sénat proposait dans le cadre de l'examen de la loi Énergie-climat, qui visait à suivre les démantèlements à venir, comme je regrette que l'ordonnance relative à l'accompagnement de la fermeture des centrales à charbon

La question de ma collègue abordait l'ensemble des aspects de la problématique sociale, économique, écologique ; ma question portera, madame la ministre, plus précisément sur l'articulation entre cette fermeture et la stratégie énergétique française dans l'optique d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le nucléaire « nous permet d'être l'un des pays qui émet le moins de CO2 pour la production d'électricité, et cela garantit notre indépendance » : ces mots ne sont pas de moi, ceux du ministre Bruno Le Maire. Ils sont frappés au coin du bon sens. Pourtant, hier, le second réacteur de Fessenheim a été déconnecté du réseau électrique Nous savons que nous ne pourrons pas réduire nos émissions de gaz à effet de serre sans décarboner notre énergie. Et nous fermons une centrale qui, justement, produit de l'électricité décarbonée Un des messages des municipales est sans ambiguïté : nos concitoyens veulent que la France se verdisse. Le meilleur vecteur est bien sûr l'efficacité énergétique. L'énergie la plus décarbonée est celle que l'on ne consomme pas Mais, à elle seule, l'efficacité énergétique ne suffira pas. Nous pouvons réviser cinquante fois la Constitution et mettre en oeuvre toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, jamais notre pays n'atteindra la neutralité carbone sans le nucléaire, malgré l'essor des renouvelables. l'oublions jamais : pour atteindre cette neutralité, il faut plus d'électricité dans notre mix énergétique et, évidemment, de l'électricité propre. En l'état actuel de la science, l'électricité renouvelable s'adosse forcément au nucléaire. Nous n'aurons donc jamais assez d'électricité renouvelable sans le nucléaire ! Madame la ministre, ne nous dites pas que l'on peut à la fois produire moins d'électricité nucléaire et décarboner moins d'énergie nucléaire, c'est forcément moins d'électricité propre, donc plus de carbone dans l'atmosphère- ce que nous aurions pu éviter de faire. Dans ces conditions, pourquoi avoir fermé Fessenheim, si ce n'est pour des raisons d'affichage ? La parole

C'est vrai, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et il est également vrai que l'énergie nucléaire est décarbonée. Mais le nucléaire, ce sont aussi des opérations de maintenance lourdes et complexes qui peuvent réduire la disponibilité du parc. C'est le cas actuellement : à la suite de la crise sanitaire, 50 % de notre parc nucléaire est aujourd'hui à l'arrêt. Je le redis : je suis convaincue de la nécessité d'un système électrique plus diversifié et plus résilient. Et puis le nucléaire, ce sont aussi des déchets. C'est donc en prenant en compte l'ensemble de ces éléments que nous avons défini la trajectoire qui figure dans la loi Énergie-climat, qui n'efface pas le nucléaire, madame la sénatrice, mais qui ramène la part du nucléaire

Cette étape est nécessaire pour garantir aux Français une production d'électricité décarbonée et résiliente. Nous avons besoin d'un meilleur équilibre entre les différentes sources d'électricité d'électricité et c'est pour cela que nous développons massivement les énergies renouvelables, que nous avons par exemple augmenté de 20 % la production d'éolien entre 2018 et 2019, que nous voulons doubler cette production dans les dix ans et multiplier par cinq la part du photovoltaïque. Je suis convaincue que c'est ainsi qu'il faut mener la transition écologique, solidaire et énergétique. Ces décisions fortes vont de pair avec un accompagnement des Français et des territoires.

Ma question s'adresse à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire. Après neuf mois de travaux, la Convention citoyenne pour le climat a présenté ses travaux, riches de nombreuses propositions. C'est bien ce qu'a souligné le Président de la République aux 150 citoyennes et citoyens réunis avant-hier à l'Élysée. Cet exercice de grande ampleur, inédit, a été largement salué un travail collectif de réflexion, de délibération, qui participe de ce nouvel élan démocratique dont notre pays a tant besoin. L'abstention, elle-même inédite, de dimanche dernier nous le rappelle si besoin.

publique -, développer les transports propres, rénover les bâtiments, investir dans l'industrie et les technologies de demain, les énergies décarbonées, les réseaux et la préservation de nos ressources en eau. milliards d'euros en plus d'ici à 2022 ont d'ailleurs été annoncés pour réussir cette transition énergétique. La quasi-totalité des mesures adoptées par la Convention devrait être reprise et trouver une traduction réglementaire lorsque cela est possible, mais aussi législative, puis référendaire. Le Président de la République a également rappelé hier que le plan de relance européen devait être nécessairement conditionné à des « engagements climatiques » de la part des États membres. C'est donc un agenda national et européen résolument tourné vers l'environnement et sa préservation se tiendra le référendum ? Pourriez-vous nous préciser, madame la ministre, l'agenda des travaux qui viendront mettre en oeuvre cette expression citoyenne ? Je pense plus particulièrement à l'agenda législatif.

le Président de la République s'est exprimé lundi sur les suites réservées aux travaux des 150 citoyens qui ont donné de leur temps personnel pour faire des propositions fortes pour le climat. Nous aussi ! Je pense que cela mérite le respect Il a fixé un cap clair et ambitieux, et montré que nous irons au bout de la transformation écologique de notre pays. D'abord, en étant au rendez-vous des attentes de la Convention, dont il a repris la quasi-totalité des propositions- 146 sur 149. Ensuite, en fixant un calendrier précis pour que cette proposition se transforme en action. Ainsi, d'ici à la fin du mois, un conseil de défense écologique assurera la mise en oeuvre des mesures qui relèvent du Gouvernement, des plans de relance- 15 milliards d'euros supplémentaires vont être consacrés à la transition écologique. Enfin, un projet de loi sera présenté à la rentrée pour les mesures qui relèvent du niveau législatif. Ce projet de loi, nous allons le construire en concertation avec les élus, les parlementaires et les citoyens de la Convention. Mon ministère, avec l'ensemble du Gouvernement, est pleinement mobilisé dans ce sens. Comme vous l'avez rappelé, agir au niveau européen est aussi essentiel. C'est pourquoi le Président de la République porte une reconstruction économique, écologique et solidaire, sur le plan national comme sur le plan européen, et les propositions de la Convention citoyenne sont au coeur de ce projet.

et Social Européen. Monsieur le ministre, il vous aura suffi d'un, lundi soir, pour terrasser le qui devait être affecté à la Lozère lors de la saison estivale, obtenu chaque année de haute lutte par les élus locaux. Il vous aura suffi d'un, lundi soir, pour rappeler un peu plus à la Lozère, département hyper-rural à l'altitude moyenne la plus haute de France, qu'il lui est si difficile d'obtenir une couverture par transport sanitaire héliporté, pourtant garantie à la quasi-totalité des territoires métropolitains à l'année. Il vous aura suffi d'un, lundi soir, pour plonger les Lozériens dans le désarroi, eux qui sont si rassurés de voir l'été leur porter assistance aux personnes ayant eu des accidents, bloquées dans des canyons ou en difficulté dans des zones inaccessibles par la route. Monsieur le ministre, en Lozère, les chances de survie lors d'un accident ou d'une maladie ne sont déjà pas les mêmes que sur le reste du territoire métropolitain. Cela est encore plus insupportable quand nos routes sont impraticables à cause des intempéries, comme c'est le cas avec la route nationale 106, seul axe routier majeur désenclavant le sud de la Lozère, fermée jusqu'à mi-juillet au moins. Alain Bertrand rappelait sur ces travées qu'il ne peut y avoir de sous-territoires ni de sous-citoyens. La Lozère ne devrait pas avoir à quémander un équipement dont les autres départements sont dotés, voire surdotés. Nous ne voulons pas, bien évidemment, priver l'Auvergne de son et encore moins entrer dans une guerre des territoires en raison de votre malheureux. Nous demandons, pour cet été, un appareil capable de remplir les mêmes missions que le, et, à terme, des engagements forts du Gouvernement pour mutualiser les appareils et permettre une couverture de notre territoire à l'année. L'égalité républicaine est un dû, pas un caprice.

Au mois de décembre, un hélicoptère de la sécurité civile a eu un accident à proximité de l'aéroport de Marignane, et je pense à ces trois personnes qui sont décédées à cette occasion.

nous pourrons immédiatement passer commande de deux nouveaux hélicoptères. Je rappelle que, la dernière fois qu'on a parlé d'hélicoptères pour la sécurité civile, il s'agissait, en 2012, de les vendre ! Et on en a vendu quelques-uns ! Depuis lors, aucun hélicoptère n'a été acheté et nous engageons cette procédure d'achat. Madame la sénatrice, ce qui compte, c'est effectivement de pouvoir garantir la sécurité de nos concitoyens, en particulier en Lozère et dans la zone concernée, pour laquelle je sais combien la montée en puissance de la saison touristique implique la présence d'un hélicoptère. Il avait été envisagé de déplacer,

affecter, cette semaine, un hélicoptère de la Gendarmerie nationale disposant des mêmes capacités d'intervention, notamment en matière d'hélitreuillage- je sais que c'est un sujet particulièrement important dans votre département -, qui sera armé par des gendarmes professionnels du secours en montagne. Cet hélicoptère sera présent, pendant les deux mois initialement prévus, prévus, sur la base de Mende. Au lieu d'un hélicoptère de la sécurité civile, ce sera un hélicoptère de la gendarmerie. Madame la sénatrice, je puis vous garantir que l'élu rural que je suis sait l'importance de ces moyens d'intervention et de cette montée en puissance pendant la saison estivale. Il y aura donc

Monsieur le ministre de l'économie et des finances, le Président de la République a pris acte des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat, dans un cérémonial quasi monarchique. Comment a-t-on pu passer d'un exercice de participation directe à une telle incarnation du pouvoir et de la décision politique ? Sur le fond, et c'est le plus important, le rejet de la proposition d'un prélèvement annuel à hauteur de 4 % sur les dividendes des grosses entreprises envoie un message politique très clair on ne touchera pas au portefeuille de ceux qui ont le plus de moyens ! Pourtant, le mouvement des gilets jaunes nous l'a bien montré : aucune justice environnementale ne sera possible sans justice sociale et, donc, sans justice fiscale. Refuser un prélèvement de 4 % des dividendes, c'est se priver de 2 milliards d'euros par an, et c'est la cohérence de l'ensemble des 149 propositions qui est remise en cause, condamnant cet exercice à une simple opération de communication malheureusement sans lendemain. Monsieur le ministre, pourquoi un tel rejet ?

En revanche, qu'il faille plus de justice fiscale, j'en suis le premier convaincu ! Qu'il faille une fiscalité plus verte, nous sommes tout à fait prêts à aller dans ce sens dans le cadre du plan de relance Mais si vous voulez une fiscalité plus juste, aidez-moi, monsieur le sénateur- et je sais que votre groupe y est prêt -, à mettre en place une taxation digitale au niveau non seulement national, mais aussi européen. Vous voulez aller chercher la richesse là où elle se trouve ? Ce sont les géants mondiaux du numérique qui ont fait les plus grands profits pendant cette crise économique ! Ce sont eux qu'il faut aller taxer et c'est cette taxation digitale qui sera juste. Vous voulez une taxation verte ? Aidez-nous à mettre en place une taxation carbone aux frontières de l'Union européenne ! En effet, rien ne sert de décarboner notre industrie française si nous ne sommes pas capables de récupérer une taxation carbone sur les produits importés de l'extérieur.

» ! Même si les élections intermédiaires sont souvent difficiles pour les gouvernements en place, celles de 2020 constituent une cuvée assez spectaculaire.

sans parler, bien sûr, des échecs de vos ministres, qui comptaient bien faire main basse sur la ville de Paris et qui, comme chacun le sait, ont eux aussi échoué. Le taux d'abstention inédit, malgré vos promesses de réconcilier les Français et la démocratie, ne relativise pas pour autant la clarté du message adressé au Président de la République et à sa majorité. Monsieur le Premier ministre, en campagne au Havre, vous avez dit aux Havrais que vous reviendriez en 2022. Ma question est simple : souhaitez-vous continuer à diriger la France, et avec quelle orientation politique ?

groupe Les Indépendants. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, la crise économique frappe le secteur automobile. Le Gouvernement a déjà annoncé un plan conjuguant relance économique et transition écologique. Malgré tout,

BorgWarner a racheté l'entreprise séculaire de Tulle en 1995, avant de transférer sa production sur une zone industrielle réalisée par le conseil départemental en 2005. Pendant plusieurs années, près de 700 salariés ont travaillé dans l'entreprise pour la fabrication de boîtes de vitesses à double embrayage, process abandonné dans les voitures électriques. La production est, à 95 %, destinée aux marques Volkswagen-Audi. Malgré les alertes réitérées des syndicats, la direction n'a pas souhaité enclencher de diversification, préparant ainsi la délocalisation de l'entreprise. Après la tristesse des employés, des familles et des responsables politiques devant cette catastrophe économique, les élus du bassin de Tulle-

devrait, dit-on, entraîner le développement de nouvelles productions ... Cette entreprise avait été créée, en 1895, pour produire des cycles.

je pourrais citer d'autres sites industriels du secteur de l'automobile, qui produisent des injecteurs diesel ou des pièces pour les véhicules thermiques -en est une illustration parfaite. Avec 368 emplois,

innovantes. La solution est-elle de préserver, à tout prix, tous les emplois liés à la production de moteurs thermiques ? Certainement pas ! C'est l'assurance d'un drame social et économique encore plus important, à une vitesse que personne ne mesure ici.

je dis bien : tout -pour trouver des solutions industrielles innovantes, permettant de garantir, non pas dans le domaine du véhicule thermique, mais sur d'autres activités, un avenir industriel à ce site de Tulle, en Corrèze.

La semaine dernière, un journal révélait que, pendant plusieurs années, les portables d'avocats de renom avaient été surveillés dans le cadre d'une enquête préliminaire ordonnée par le parquet national financier Cette enquête, décidée pour une prétendue violation du secret professionnel, a été ordonnée alors que, quelques jours avant, le 26 février 2014, une information judiciaire avait été ouverte sur des faits connexes. Malgré l'absence de preuves, le parquet national financier l'a relancée en octobre 2016, sans succès non plus. En décembre 2019, un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » est même prononcé. Les conditions de cette enquête sont troublantes. Elle n'a pas été jointe au reste de la procédure pendant longtemps et ses résultats ont été cachés à la défense. Le PNF a agi comme une juridiction d'exception, qui nous rappelle les pires errements d'une justice livrée à elle-même. L'autorité judiciaire ne saurait être hors contrôle Veiller à l'intégrité des comptes publics ou privés est une chose ; régler des comptes avec les hommes politiques en est une autre ! « La cour rend des arrêts, et non pas des services », disait un grand magistrat du XIX siècle. du parquet national financier dans le jeu politique nous a même valu, voilà trois ans, une élection présidentielle insolite, où le favori n'a même pas été qualifié pour le second tour. À la suite de propos tenus par l'ancienne procureure du PNF, le Président de la République a saisi le Conseil supérieur de la magistrature et vous, madame la garde des sceaux, avez demandé timidement un rapport circonstancié sur la nature précise de l'enquête qui Il était temps de saisir l'inspection générale de la justice, car c'est l'existence même du PNF qui pose problème. Madame la garde des sceaux, qu'entendez-vous faire face à cette crise de confiance envers la justice, pour que, après le « mur des cons », ne s'érige pas le « mur de la honte »

je comprends l'émotion qu'ont suscitée les propos de Mme Éliane Houlette, lors de son audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez rappelé, le Président de la République, qui est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, a sollicité un avis du Conseil supérieur de la magistrature.

-un rapport à Mme la procureure générale de Paris, qui me l'a rendu hier soir. À la lecture de ce rapport, j'ai immédiatement décidé de saisir l'inspection générale de la justice, afin que celle-ci puisse déterminer

La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour le groupe socialiste et républicain. Le Président de la République recevait lundi les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Notre groupe tient à saluer la qualité des travaux menés par ce panel de citoyens, qui se sont engagés en faveur d'une transition écologique ambitieuse pour notre pays. Le chef de l'État a indiqué reprendre 146 des 149 propositions formulées et souhaiter les transmettre « sans filtre » au Parlement pour ce qui relève de la loi. Un texte comprenant diverses mesures est ainsi annoncé pour la rentrée. Nous aurions besoin d'éclaircissements sur ce point et, surtout, de l'assurance que ces mesures seront bien accompagnées des financements nécessaires sur le court terme, et pas seulement dans un cadre pluriannuel. Sur le sujet, par exemple, de l'agriculture et de l'alimentation durables, qui me tient particulièrement à coeur, les enjeux économiques sont effectivement indissociables des enjeux environnementaux. Il faut renforcer la lutte contre les inégalités sociales face à l'alimentation les agriculteurs doivent être accompagnés dans la transition agroécologique en termes d'aide financière, mais aussi de formation. Sans engagement résolu de l'État en la matière, les propositions formulées risquent de rester lettre morte.

Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous agir ? Il est encore temps d'éviter ce genre de désastres, dans des territoires en difficulté, et d'être véritablement en cohérence avec les engagements de la Convention citoyenne pour le

durant laquelle tous nos soignants ont été au front, jour et nuit, que vous les aviez enfin entendus et que les problèmes les plus urgents, notamment les dégradations des conditions de travail et les rémunérations insuffisantes, allaient être pris en considération. Or il n'en est toujours rien aujourd'hui ! Le Ségur de la santé ne répond pas aux questions, car nos soignants sont de nouveau dans la rue. Ces mêmes soignants qui ont risqué, parfois perdu la vie pour nous sortir de la covid-19. Ces mêmes soignants que nous applaudissions tous les soirs à la même heure pour les remercier de leur dévouement et de leur engagement. Ces mêmes soignants qui sont en droit d'attendre mieux, et plus, que des médailles ou quelques primes. Les faits et les chiffres sont là. En France, nos médecins hospitaliers sont payés 40 % de moins que leurs collègues allemands. Nos infirmiers, comme nos aides-soignants sont rémunérés 20 % de moins que leurs homologues européens. Mais cela va encore plus loin : l'administration a submergé la santé en France, tout particulièrement l'hôpital, où le personnel soignant et sachant a depuis longtemps perdu tout pouvoir. Oui, nous l'affirmons, notre système de santé actuel est d'abord malade de la sur-administration ! Il y a urgence à repenser toute l'organisation du travail des services publics de santé les charges administratives ne doivent plus entacher leur quotidien ; la gouvernance des hôpitaux doit être reconsidérée ; les moyens humains et logistiques adaptés ; le management et la formation améliorés. Le Gouvernement va me répondre qu'il vient, au travers du Ségur de la santé, d'annoncer des revalorisations. Ces dernières ne répondent pas aux attentes légitimes des professionnels de santé, qui n'ont pas de mots assez forts pour critiquer ce qui n'est toujours que du saupoudrage. Pourquoi le Ségur de la santé élude-t-il les problèmes de gouvernance à l'hôpital ? Pourquoi renoncer à « dégraisser le mammouth administratif »

Dans le cadre du Ségur de la santé, nous discutons également d'un nouveau plan d'investissement pour les établissements de santé, les Ehpad et le numérique en santé. Le troisième est le travail sur le

Cette rencontre avait permis d'établir deux objectifs pour gagner cette guerre : d'abord, combattre les terroristes ; ensuite, former et équiper les armées nationales. N'oublions jamais que, chaque jour, nos soldats livrent un âpre combat contre les djihadistes dans le Sahel.

La mobilisation européenne à nos côtés se confirme, même si elle reste encore trop lente. La Takuba est, à cet égard, aussi importante que représentative. Madame la ministre, l'Estonie sera-t-elle le seul pays européen à nous rejoindre ? Mais, après avoir gagné la guerre, le plus dur est souvent de gagner la paix. Vous l'avez dit vous-même, une opération telle que Barkhane n'a pas vocation à être pérenne. L'action militaire est, non pas une fin en soi, mais un moyen au service d'un objectif global, qui a motivé notre présence permettre à des États de demeurer libres et de fonctionner normalement, de manière indépendante, au service de leur population. C'est pourquoi deux objectifs avaient été fixés à Pau pour gagner la paix : le retour des États dans les territoires ravagés par le djihadisme et l'aide au développement de la région. Toutefois, le Président de la République l'a admis lui-même à son arrivée à Nouakchott, hier, il faut en faire davantage dans ce domaine. Ma question est donc simple : où en est l'Alliance Sahel et sommes-nous sur la bonne voie ? La parole

Cela nous a permis, tous ensemble, d'engranger des succès, notamment militaires, et de donner un nouvel élan à notre action. Ce nouvel élan, c'est celui de la coopération. Au Sahel, la victoire est effectivement possible si nous restons unis, si nous unissons nos forces avec les pays du G5 Sahel et avec les Européens. Il faut le faire pour accompagner au combat les forces armées locales. ces forces armées sahéliennes est visible. Des camps militaires ont été repris et le niveau de coopération s'est grandement amélioré.

À cet égard, l'action militaire n'est effectivement pas une fin en soi : il faut pouvoir aider les pays du Sahel à faire face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux. C'est pourquoi, sur le terrain, les militaires de l'opération Barkhane continuent d'accompagner le retour de l'État, comme ils l'ont fait encore récemment à Labbezanga- eh oui, les populations reviennent ! Bien sûr, il faudra faire plus, mais les premiers signaux sont là. Nous sommes sur la bonne voie

Deromedi, pour le groupe Les Républicains. Les conséquences de la double crise sanitaire et économique affectent considérablement un grand nombre de Français résidant hors de France. Le 30 avril dernier nous a été présenté un dispositif de soutien aux Français de l'étranger de 220 millions d'euros, auxquels viennent de s'ajouter 35 millions d'euros. C'est mieux, mais cela reste malheureusement très insuffisant ! J'ai conscience de la difficulté d'ouvrir, sur le budget de l'État, des aides aux Français de l'étranger, mais nous n'avons pas le choix. La France n'a pas le droit d'abandonner ses enfants, où qu'ils soient. Il s'agit là d'un appel au secours de personnes qui n'ont jamais tendu la main, mais qu'il faut soutenir pour quelques mois. Il faut un plan d'urgence à la hauteur de la situation Il doit inclure, outre l'aide sociale et le soutien à l'enseignement français, le soutien aux entrepreneurs. Certains d'entre eux connaissent de graves difficultés financières, en particulier dans les secteurs impactés directement par la crise. Ils contribuent aussi au développement économique de la France, mais ne bénéficient pas, la plupart du temps, d'aides dans leur pays d'accueil. Comment le Gouvernement accueillera-t-il les familles ou les retraités qui n'arrivent plus à vivre à l'étranger, ceux que les familles ne peuvent pas prendre en charge

4 tonnes de médicaments ont été préacheminées pour faire face à d'éventuelles ruptures de stocks dans le système commercial local et un système d'évacuation sanitaire, reposant sur 3 avions,

Les Français résidant hors de France ne souhaitent pas rentrer, si vous leur donnez la possibilité de rester dans leur pays d'accueil. Il s'agit de les aider pour quelques mois. Ou bien il faudra les rapatrier, dans des conditions qui ne feront pas honneur à la cinquième puissance mondiale

ils sont, pour nos territoires et nos concitoyens qui y vivent, source de lien social et de richesse. De fait, nos commerces sont des lieux d'échanges qui contribuent à l'attractivité et au dynamisme de nos communes. En étant au plus près des attentes de nos concitoyens et en leur offrant des produits et services de qualité, ils sont, en quelque sorte, l'âme de nos territoires. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre, nos commerçants, artisans et indépendants souffrent. Ils souffrent car, du fait de la crise sanitaire qui frappe notre pays, bon nombre d'entre eux ont été privés de toute activité durant près de trois mois. Malgré les aides dont ils ont bénéficié, nombre d'entre eux craignent de ne pas pouvoir se relever, d'autant qu'ils étaient déjà fragilisés par la crise des gilets jaunes et les autres mouvements sociaux que nous avons récemment connus. Ils souffrent car, nous le savons, l'activité économique est bien loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant-crise, et le retour à la normale sera très long. vous avez annoncé, monsieur le ministre, un plan de soutien à hauteur de 900 millions d'euros pour aider les commerçants, artisans et indépendants. Ce plan prolonge les dispositifs existants, notamment l'activité partielle, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État et le report des charges fiscales et sociales. et sociales. Destiné à renforcer leur trésorerie, il constitue une réponse concrète aux attentes de nos commerçants, artisans et indépendants, dont le chiffre d'affaires a déjà considérablement baissé. La redynamisation du commerce de proximité est une exigence pour nos centres-villes et centres-bourgs, chère à Rémy Pointereau et Martial Bourquin ; gage d'attractivité pour nos territoires, elle est une véritable richesse pour nos concitoyens qui y vivent. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous fournir plus de précisions sur ce plan, qui permettra, je l'espère, de répondre à un secteur

artisans et indépendants sont, probablement, ceux qui ont le plus souffert de ces mois de crise. Tout simplement parce qu'ils étaient fermés et qu'ils ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 50 %, 60 %, parfois 80 %, sans aucune solution disponible. raison pour laquelle le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics et moi-même avons déployé toute une série d'instruments très puissants : le fonds de solidarité, les exonérations ou reports de charges sociales et fiscales, le chômage partiel, toutes mesures qui leur ont permis de passer ces quatre mois de crise avec le moins de dégâts possible. Maintenant, nous voulons faire plus. Nous voulons faire plus pour revitaliser un certain nombre de centres-bourgs et de centres-villes, et pour aider les commerçants, indépendants et artisans dans les mois qui viennent.

totalement nouveau, efficace et qui permettra de voir des commerces rouvrir dans les centres-villes et les communes rurales. Enfin, nous allons engager un plan de numérisation et de digitalisation de tous les commerces. En effet, la crise a montré que ceux qui sont digitalisés s'en sortent le mieux. Vous le voyez, nous avons fait beaucoup. Nous ferons davantage encore pour les indépendants et les commerçants

Hier, à Paris, la police a procédé à des contrôles d'identité. Tout s'est bien passé : les citoyens avaient leur document d'identité, ils n'étaient ni arrogants ni irrespectueux, ils n'ont pas tenté de fuir, aucun d'entre eux n'était recherché, il n'y eut aucune esclandre et les policiers n'ont pas été filmés ni insultés ; ceux-ci ont été courtois et polis, comme ils le sont toujours dans l'exercice de leurs nombreuses missions au contact. Bravo ! Pourtant,

leur moral est au plus bas. Nos policiers se sentent abandonnés, peu soutenus, ni écoutés ni compris. Bref, ils sont en grande souffrance. Nous Nous n'avons cessé de le souligner avec force ces trois dernières années dans nos rapports sénatoriaux sur les programmes 176 et 152 des projets de loi de finances, issus des commissions des finances et des lois, surtout dans le rapport de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité, que nous vous avons remis à la fin de 2018. Tout y est dit ! Sans résultats concrets en réponse ... Alors que notre édifice sécuritaire craque de toutes parts, parts, monsieur le Premier ministre, nos forces de l'ordre continuent à accomplir un travail constant remarquable, tout en étant à bout de souffle- et ce n'est pas, loin de là, un mouvement d'humeur. Lorsque l'un des piliers de l'ordre vacille, la santé de la République est bien en danger ! Ma question est donc simple, très simple : après le Ségur de la santé, à quand le Beauvau de la sécurité ? Le livre blanc annoncé est déjà obsolète ...

est la réalité à laquelle nous devons faire face. Le Livre blanc de la sécurité intérieure doit permettre, à partir de l'ensemble des constats, de définir une nouvelle sécurité, à hauteur d'hommes

! La parole est à Mme Marie-Noëlle Schoeller, pour le groupe socialiste et républicain. Je salue sa première prise de parole dans notre hémicycle parole dans notre hémicycle ! Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le ministre, en 2003, le pays mesurait la part, le poids et la gravité de l'isolement dans la surmortalité de nos anciens. Il y eut un plan canicule. En 2020, la pandémie induit des mesures drastiques de sécurité sanitaire : nos aînés sont, où qu'ils soient, isolés et même mis sous cloche. S'il était impératif de les protéger, comme les soignants, d'un virus pernicieux, convenait-il de le faire au détriment de toute humanité, au point d'oublier les enseignements de 2003 ? Dans les structures médico-sociales, dès le 7 mars, il n'y a plus eu ni visites, ni journaux, ni livres, ni animations partagées, ni repas en commun ; la kinésithérapie a été réduite, les vêtements personnels parfois retirés. Reste le téléphone, pour qui n'est pas sourd, et Skype, s'il est du personnel pour assurer les liaisons ... En ville, l'aide à domicile se concentre sur les plus dépendants. Pour les autres, la solitude devient abandon : plus d'aide-ménagère, de visites, de kiné. Les accueils de jour sont fermés : tout s'arrête, et les repas sont déposés sur le seuil de la porte. Tous les personnels ont fait le maximum pour que, en l'absence des familles, nos anciens soient entourés- sans protection d'abord, car oubliés du système, et sans les nécessaires renforts de personnel. le coût humain est lourd : privés, sans le comprendre, de la présence de leurs proches, certains se sont laissés mourir de chagrin et d'ennui ; d'autres subissent des pertes irréversibles d'autonomie, sur le plan de la motricité- faute d'entraînement physique -ou de la mémoire- faute de repères et de stimulation. De vieux couples ont attendu trois mois pour se voir. Des familles ont eu la douleur d'enterrer leur mort à la sauvette, sans un dernier regard ... Monsieur le ministre, envisagez-vous d'établir pour l'avenir un plan Pandémie qui prenne mieux en compte les aînés et leurs proches ? La parole

le report des élections régionales est à l'ordre du jour, on parle assez peu des élections départementales. Or, afin de lutter contre l'abstention, un consensus se dégage depuis de nombreuses années pour regrouper les élections locales ce fut d'ailleurs l'objet de la loi de 2015. Dans ces conditions, monsieur le ministre, l'éventuel report des élections régionales serait-il couplé avec un report identique des élections départementales ?

politique, vous le connaissez. Il s'agit de faire en sorte que toute la France soit totalement tournée vers un seul objectif : la reconstruction économique et sociale de notre pays. Pour cela, nous avons besoin de nous appuyer sur des collectivités territoriales puissantes, notamment pour réaliser la reconstruction économique.

C'est la raison pour laquelle une réflexion- je dis bien : une réflexion -a été engagée sur cette ambition que nous devons construire tous ensemble, y compris, évidemment, avec les sénateurs, pour se projeter vers l'avenir d'une réorganisation institutionnelle dont notre pays a besoin. S'agissant de votre question précise, monsieur le sénateur, s'il y avait,

La séance est reprise. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- quinze voix pour, une voix contre -à la nomination de M. Jean-Philippe Vachia aux fonctions de président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. L'ordre du jour appelle la désignation des trente-six membres de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion. En application de l'article 8, alinéa 5, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion commune du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la dette sociale et à l'autonomie J'informe le Sénat que les candidatures pour siéger au sein des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer les textes sur les dispositions restant en discussion de ces projets de loi ont été publiées.

C'est ce que permettent ces deux textes, dans des circonstances certes particulières, il faut le reconnaître. Cette nouvelle reprise de dette par la Cades est une nécessité de court terme au regard de la situation que nous traversons et qui nous inquiète tous ; mais c'est aussi un outil nous permettant de regarder en face les grands défis de notre temps.

Il y a quelques mois, le retour à l'équilibre des comptes sociaux était proche, et nous débattions pour savoir à quel moment de l'année 2024 la dette sociale reprise par la Cades arriverait à échéance. La crise sanitaire, devenue crise économique, rebat désormais les cartes. Nous assistons à la reconstitution de déficits importants. Nous le regrettons tous, évidemment, mais c'est aussi le prix à payer d'une politique extrêmement volontariste, de la part du Gouvernement, pour faire face à la crise : la protection dont ont bénéficié les Français a peut-être été la

Même dans la perspective d'un rebond de l'économie, que nous attendons tous et auquel nous travaillons, les déficits sont inéluctables. En conséquence, seul un transfert important peut permettre à la Cades des placements à horizon long, qui sont les plus sécurisants et seule cette reprise nous protégera contre le risque de devoir décaler un jour le paiement des prestations, faute de financement. Avec ce projet de loi, nous proposons donc une opération de bonne gestion de la sécurité sociale nous renouvelons l'engagement de rembourser les dettes de la sécurité sociale, dont une partie découle de la crise actuelle. Agir ainsi, c'est respecter les principes de 1996, selon lesquels la dette sociale est gérée vertueusement et apurée au principal. Concrètement, cela signifie que nous devons prolonger la durée pendant laquelle nous mobilisons des recettes pour rembourser la dette pour neuf années supplémentaires, de 2024 à 2033. Je devance sans doute une partie des débats en formulant ce rappel : le Gouvernement tient à ce que cette reprise de dette sociale inclue 13 milliards d'euros pour les hôpitaux. le déficit de l'assurance maladie et celui de nos hôpitaux sont liés : les économies de la première ne peuvent se transformer en déficit pour les seconds. En supprimant cette reprise, la commission prive ainsi les hôpitaux d'une bouffée d'air. Or ce financement

En 1945, il a été décidé de créer une assurance sociale publique contre le risque de maladie ou d'accident du travail : nous faisons aujourd'hui le choix d'une nouvelle assurance publique, contre ce qui est devenu un nouveau risque, auquel tous les Français peuvent être

Dès lors, je l'ai indiqué à la commission, il est temps de se poser les mêmes questions fondamentales qu'en 1996. Est-il nécessaire d'amortir la dette sociale ? Est-ce possible ? Le cas échéant, comment faire pour y parvenir ? À l'inverse, ne serait-il pas préférable d'employer dès à présent à un autre usage les moyens dédiés à l'amortissement de cette dette ? Dans sa majorité, la commission a considéré que nous devions conserver pour objectif l'extinction totale de cette dette. En effet, la sécurité sociale est fondamentalement un système d'assurance sociale et de répartition. Par nature, les dépenses de sécurité sociale ne sont pas, comme certaines dépenses de l'État, un investissement dont bénéficieront les Français de demain

La logique d'une poursuite de l'équilibre des comptes sociaux n'est pas une obsession de comptable : c'est fondamentalement une affaire de solidarité entre générations. C'est pour cela que nous devons sortir de cette histoire apparemment sans fin, en nous donnant les moyens d'y parvenir, à la date fixée et selon les objectifs définis. deux conditions nous ont paru nécessaires : d'une part, s'assurer que la dette transférée à la Cades est bien légitime ; d'autre part, couper, quand ce sera possible, le robinet des déficits de la sécurité sociale, qui alimente les futurs transferts de dette sociale. S'agissant de la légitimité de la dette transférée, la commission a approuvé le transfert des dettes passées des différents régimes de sécurité sociale : elle en souligne la nécessité depuis plusieurs années déjà. Elle a également adopté le transfert des déficits prévus pour les exercices 2020 à 2023, en espérant qu'ils soient inférieurs aux 92 milliards d'euros provisionnés. À cet égard, la part conjoncturelle de ces déficits constitue bien de la dette sociale. En revanche,

Comme l'ont souligné la Cour des comptes, puis, plus récemment, l'IGF et l'IGAS, comme beaucoup d'entre nous ont pu le voir en exerçant un mandat local, cette dette est très largement due à des investissements immobiliers surdimensionnés ou, en tout cas, mal maîtrisés, réalisés sur l'initiative de l'État et sous la tutelle parfois défaillante du même État, notamment dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012. Dans ces conditions,

Il est ainsi proposé que le cumul des soldes consolidés des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV des années à +4 soit toujours positif ou nul

en léguant le coût à nos enfants. Elle est souple, parce que, dans ce cadre, les déficits ponctuels resteront permis, l'équilibre étant constamment apprécié sur un moyen terme, celui d'un cycle économique. De plus, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles comme celles que nous vivons, l'échéance pour retrouver un équilibre global pourrait être étendue jusqu'à dix ans. dix ans. Je serai beaucoup plus bref pour ce qui concerne le volet « autonomie » des deux textes, non du fait de son importance, qui est grande, mais parce que la commission ne l'a que peu amendé par rapport au texte de l'Assemblée nationale.

N'est-il pas étrange de demander un rapport « fondateur » au Gouvernement et d'en anticiper toutes les conclusions, notamment en termes d'organisation et de financement ? En outre- je m'adresse directement à vous, monsieur le secrétaire d'État -, quelle serait la place, dans le cadre de cette branche, des différentes parties prenantes dans le secteur de l'autonomie,

à ce que l'élaboration du rapport du Gouvernement associe toutes les parties prenantes, notamment les différents acteurs du grand âge et du handicap, les collectivités territoriales et les aidants. Enfin, soyons conscients que le plus dur reste à faire. faire. Au fond, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nouveaux moyens financiers, comme l'a souligné le rapport Libault, et d'une nouvelle culture de la prise en charge du grand âge. Il faut revoir l'organisation de la prise en charge de l'autonomie. L'Ehpad ne doit plus en être l'alpha et surtout l'oméga,

sont destinés à répondre à une urgence : la crise sanitaire, qui est venue grever les comptes des régimes sociaux. Finalement, les trois séries de remarques que je vais développer ci-après viennent illustrer l'adage : « Vite et bien ne s'accordent guère.

par la sécurité sociale. En effet, sur les 136 milliards d'euros de dette transférés, 50 milliards d'euros relèvent de la pandémie de covid, mais certains coûts inclus dans cette enveloppe ne sont pas des dépenses d'assurance maladie. Je citerai, par exemple, la fourniture de dispositifs médicaux pour le personnel soignant ou encore la revalorisation des traitements. Quant à la dette des hôpitaux, elle relève avant tout d'une logique d'investissement immobilier.

précédés. L'allongement de la durée de vie met également en cause la diminution des prélèvements obligatoires, attendue à partir de 2024 avec la disparition de la CRDS.

je le dis pour l'information de tous -, la commission des finances ne pouvait manquer de souligner que l'affectation à une dépense nouvelle d'une ressource initialement dédiée à l'apurement d'une dette va dégrader, au sens de la comptabilité nationale et des critères de Maastricht, le solde public.

dans un sens très large, ne va pas conduire au gel de toute réforme quant au financement des régimes sociaux. En 2018, c'est uniquement un retournement de conjoncture qui a laissé entrevoir un rapide retour à l'équilibre.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis trente ans, les gouvernements successifs soutenus par le patronat n'ont eu de cesse de stigmatiser le « trou abyssal de la dette de la sécurité sociale Cette dette, sciemment entretenue, quelle est-elle et surtout d'où vient-elle ? La dette sociale est le résultat des politiques de diminution des ressources de la sécurité sociale davantage que de l'augmentation des dépenses. La crise du covid-19 a entraîné une augmentation des dépenses publiques, avec la prise en charge de l'activité partielle pour les entreprises, les reports de charges financières et les exonérations de cotisations sociales. Cette dette correspond en réalité au coût des décisions prises par le Gouvernement durant l'épidémie de covid-19 et à ses conséquences pour les années à venir. Plutôt que d'en assumer la responsabilité, le Gouvernement a préféré transférer la facture des politiques publiques au budget de la sécurité sociale. Pour le dire autrement, l'État, qui pioche déjà chaque année dans le porte-monnaie de la sécu, a décidé d'inscrire directement en haut de la facture du covid-19 le nom de la sécurité sociale. Non seulement un tel procédé contrevient à la répartition des missions régaliennes et de la sécurité sociale, mais ce transfert de dette est une mauvaise opération comptable. Le Gouvernement aurait pu faire assumer la dette sociale par l'État par l'État : il s'agit d'une dette exceptionnelle résultant, non pas d'une mauvaise gestion de la sécurité sociale, mais de décisions prises par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire. La prise en charge par l'État de la « dette covid » serait une meilleure opération sur le plan financier, puisque la dette de l'État est gérée à très long terme à un taux avantageux. À l'inverse, la Cades rembourse les déficits cumulés par les organismes de sécurité sociale à moyen terme et dans des conditions moins avantageuses. Ainsi, selon l'économiste Michaël Zemmour, si l'État prend en charge la « dette covid », il lui en coûtera de l'ordre de 1 milliard d'euros par an, et cette dette pourra être gérée comme une dette exceptionnelle appuyée par la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Or le Gouvernement préfère transférer à la Caisse d'amortissement de la dette sociale une dette de 136 milliards d'euros, dont 31 milliards d'euros viennent de la reprise de déficits passés

a tant mélangé les circuits de financement entre l'État et la sécurité sociale, en compensant les exonérations de cotisations par des ponctions de TVA, que les parois des deux budgets ne sont plus étanches. Le Gouvernement utilise la confusion des dépenses sociales pour faire discrètement payer à la sécurité sociale les décisions prises durant la crise du covid-19. Pourtant, la « dette covid » concerne toute la Nation. En ce sens, elle doit être gérée par l'État. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : le Haut Conseil du financement de la protection sociale et la Fédération hospitalière de France suggèrent que l'État assume cette dette dans un dispositif spécifique à long terme. Le projet de loi organique remet en cause l'autonomie financière de la sécurité sociale, l'autonomie de sa gouvernance, l'autonomie de son mode de fonctionnement et enfin l'autonomie de son mode de financement. Le Gouvernement remet Le Gouvernement remet en cause l'autonomie financière de la sécurité sociale en refusant de compenser les pertes de recettes dues aux exonérations de cotisations sociales des entreprises qu'il a lui-même Ainsi, ce sont 30 milliards d'euros de pertes de recettes, qui, du fait des reports de cotisations et contributions sociales, sont transférés à la sécurité sociale.

Enfin, 8 milliards d'euros de l'assurance maladie sont transférés, alors qu'il s'agit du budget de l'agence Santé publique France pour reconstituer ses stocks stratégiques, du versement de primes au personnel des établissements publics de santé comme des Ehpad et de l'augmentation des indemnités journalières, étendues aux personnes contraintes de garder leurs enfants. En résumé, l'autonomie financière de la sécurité sociale est remise en cause après le transfert d'une dette dont près de la moitié devrait être affectée au budget de l'État. La droite sénatoriale est allée plus loin dans la logique uniquement comptable de la sécurité sociale, car, sous prétexte de préserver les équilibres de la sécurité sociale, elle a proposé d'inscrire dans la loi organique une « règle d'or Cette règle d'or est la même qui justifie au niveau européen les politiques d'austérité depuis trente ans. Avec votre règle d'or, les futures lois de financement de la sécurité sociale ne seront plus autorisées à alimenter la Cades par de nouveaux déficits. pensez ainsi supprimer les déficits en les interdisant, un raisonnement simpliste qui va à contre-courant de la crise qui vient de se produire et qui devrait nous conduire à davantage de modestie en matière de certitudes économiques. En réalité, votre objectif est d'inscrire l'austérité dans le marbre, alors que les personnels hospitaliers demandent actuellement que les hôpitaux soient enfin financés à la hauteur des besoins. C'est vous qui serez responsables, demain, des lits supprimés et des services fermés avec votre règle d'or Ce projet de loi est dangereux, car il remet en cause l'autonomie de la gouvernance de la sécurité sociale. En effet, cette réforme n'a pas été présentée devant l'ensemble des instances de la sécurité sociale. Alors que nous examinons ces deux projets de loi, la commission des comptes de la sécurité sociale n'a pas encore été saisie, et le Haut Conseil du financement de la protection sociale a rendu un avis contraire.

En effet, la création de la nouvelle branche de la sécurité sociale que vous prévoyez serait assurée par le financement exclusif des assurés sociaux- travailleurs, chômeurs ou ayants droit -, sans aucune participation financière des employeurs. notre système trouve ses fondements dans son financement à partir de la cotisation sociale, qui est la part socialisée du salaire mutualisé entre les salariés.

patronales, la part des cotisations sociales dans le budget de la sécurité sociale ne représentait plus que 50,7 % des recettes Nous assistons donc à une étatisation forcée de la sécurité sociale, qui devient une variable d'ajustement du budget de l'État, le social étant mis à contribution des orientations austéritaires du libéralisme européen. Il faut dire qu'agiter le « trou de la sécurité sociale » permet de justifier la baisse des prestations et de préparer le terrain pour réduire les pensions de retraite lors de la future réforme ! La seconde partie de ce projet de loi concerne la perte d'autonomie.

Il s'agit donc d'un coup de communication du Gouvernement, qui a mis la charrue devant les boeufs. Le rapport Libault de mars 2019 prônait la création d'un cinquième risque, mais s'opposait à la création d'une cinquième branche, considérant que confier sa gestion à une branche de sécurité sociale « impliquerait l'effacement du département et le transfert de la gestion des prestations à un des réseaux existants de caisses locales ».

intégré dans un grand service public de santé et de l'action sociale, dont le financement serait assuré par l'arrêt des exonérations de cotisations sociales

Je rappelle que les services d'aide à domicile ont été exemplaires durant cette crise, alors que les personnels connaissent des conditions de travail extrêmement difficiles et pénibles ainsi qu'une faible rémunération. Le Gouvernement a renvoyé aux départements la responsabilité d'assurer le paiement d'une prime aux personnels de l'aide à domicile, alors que les dotations aux collectivités ont diminué de 30 milliards d'euros en 2020. Avec votre projet de loi, vous bafouez le principe d'autonomie organique et financière reconnu par notre législation républicaine, je veux parler notamment de l'article 13

Le scrutin est ouvert.

à constater le résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,

qui, dans son discours solennel du 14 juin dernier- il y a quinze jours -, annonçait que la France ne financerait pas les dépenses de la crise sanitaire en augmentant les impôts. Mes chers collègues, force est de constater que transférer à la Cades 136 milliards d'euros de dette

Et pas n'importe quel impôt : un impôt particulièrement injuste, puisqu'il ponctionne l'intégralité des salaires sans aucune progressivité ! Et pas n'importe quand : l'impôt créé sera appliqué entre 2024 et 2033, c'est-à-dire intégralement après la présente mandature, ce qui n'est pas sans poser une question démocratique ! Il vous faut désormais l'assumer, monsieur le secrétaire d'État : plutôt que de rétablir l'impôt sur la fortune, de solliciter les plus aisés, le capital, les dividendes, vous avez décidé de créer un impôt qui, en pratique, va pénaliser davantage les plus modestes. Au-delà même de cette décision injuste, nous trouvons la logique de transfert de dette aux comptes sociaux très contestable en termes de gestion. En effet, cette décision va grever nos comptes sociaux,

la dette que vous avez décidé de réduire les droits des chômeurs et des plus précaires. Aujourd'hui, la dette de l'État est transférée. Or cette dette exceptionnelle résulte majoritairement de choix politiques visant à répondre à un événement lui-même exceptionnel et mondial. Elle

nous persistons à penser que la sécurité sociale doit financer les dépenses sociales et qu'on ne doit pas lui faire porter les choix politiques du Gouvernement. Mes chers collègues, à quoi correspondent ces 136 milliards d'euros de dette que le Gouvernement entend transférer à la Cades ?

si l'État prend en charge cette " dette covid ", il lui en coûtera de l'ordre de 1 milliard d'euros par an [ ...], et cette dette pourra être gérée comme une dette exceptionnelle, appuyé en cela par la politique monétaire non conventionnelle de la Banque centrale européenne.

fois- nous n'en sommes plus surpris -, entraînent la baisse des droits pour les plus fragiles. Vous souhaitez mettre la pression sur les dépenses de protection sociale

: il vous a été utile de communiquer sur la mise en oeuvre d'une telle réforme pour faire passer la pilule de la dette sociale ! À la lecture de l'intitulé du projet de loi, nous avons tous cru qu'enfin le cinquième risque, que nous appelons de nos voeux depuis plusieurs années avec les associations, les familles et les départements, allait être mis en oeuvre. En réalité,

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

mon sentiment de perplexité devant une séquence législative qui, au hasard d'un amendement sur une proposition de remise d'un rapport et la mise en place en 2024 d'une dérivation de tuyauterie de CSG, nous conduira à approuver ou refuser en même temps la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale- rien que cela ! -et le traitement de 136 milliards d'euros

la définition des prestations qui transformeront- peut-être -la secousse médiatique en événement historique dans l'histoire de la sécurité sociale. J'affirmerai pour ma part notre opposition au transfert de 136 milliards d'euros à la Cades, correspondant à une reprise de dettes passées, de dettes en cours de constitution et même futures, auxquelles s'ajoutent, hors de tout lien avec les missions de la Cades, 13 milliards d'euros de dette hospitalière. désaccord avec des décisions financières qui relèvent de choix politiques fondamentaux quant à la philosophie de la sécurité sociale. L'autonomie est un pilier fondateur de celle-ci, conforté par la loi Veil de juillet 1994. la création de la CSG et l'évolution vers le caractère universel ont bousculé les principes de 1945, mais, surtout, monsieur le secrétaire d'État, vous avez, ces dernières années, par la suppression de cotisations et par la non-compensation d'exonérations, accentué la confusion entre les périmètres de la protection sociale et du budget de l'État. Au moment où un événement mondial sans précédent affecte la santé publique, multiplie situations précaires et pauvreté, augmente le chômage, met en danger des pans entiers de notre économie, vous réaffirmez la stricte autonomie de la dette sociale et vous portez à la charge des assurés sociaux des milliards de dettes non liées à leurs comportements ou à une mauvaise gestion des caisses- c'est un deuxième point d'incompréhension. La sécurité sociale ne peut pas être autonome quand elle est en déficit et ne plus l'être quand des excédents sont espérés.

Les décisions de la BCE garantissent certainement des taux très bas pour les dix ans à venir. Surtout, on libérerait ainsi, et sans conséquence pour le budget de l'État, une source de recettes de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros chaque année, qui permettrait de construire enfin un nouvel équilibre réel de la sécurité sociale, prenant en compte les besoins des hôpitaux, les nouvelles thérapies et la création tellement attendue d'une cinquième branche.

Quel plaisir de retrouver l'hémicycle et de vous retrouver, mes chers collègues, après trois mois d'absence ! Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'ampleur inédite de la crise sanitaire qui nous frappe a fortement impacté les finances sociales et a mis notre système de sécurité sociale à rude épreuve. Au début du mois de juin, le ministre de l'action et des comptes publics estimait que le déficit de la sécurité sociale s'établirait à 52,2 milliards d'euros en 2020, contre une prévision initiale de 5,4 milliards Il est donc dix fois plus important que prévu. Afin de répondre à l'aggravation du déficit, le Gouvernement nous présente ces projets de loi, qui visent deux objectifs : transférer une partie de la dette à la Cades et créer une cinquième branche de la sécurité sociale relative à l'autonomie. le transfert de la dette, dans l'ensemble, les coûts considérables engendrés par l'épidémie de covid-19 résultent notamment de la contraction de la masse salariale du secteur privé, des reports de cotisations accordés aux entreprises pour soulager leur trésorerie, des dépenses pour combattre la propagation du virus et rémunérer les personnels hospitaliers. Si ces sommes colossales vont peser sur les finances publiques, elles n'en étaient pas moins nécessaires. Elles sont la résultante de mesures d'urgence, qui ont été prises en période de crise et que l'État se doit d'assumer.

Cades. Ce choix peut prêter à débat, mais est somme toute logique, puisque l'objectif de la Cades est d'apurer les déficits de la sécurité sociale, que la crise a aggravés. En revanche, parmi les 136 milliards d'euros transférés figurent les 13 milliards d'euros de dette des hôpitaux que le Gouvernement, par la voix de Mme Agnès Buzyn, s'était pourtant engagé, au nom de l'État, à reprendre en novembre dernier. Ce transfert ne me paraît donc pas justifié. Aussi, je me félicite que la commission des affaires sociales ait suivi la proposition de notre rapporteur de supprimer la reprise de la dette des hôpitaux par la Cades. Comme l'a rappelé notre président Alain Milon, les hôpitaux appartiennent à l'État et non à l'assurance maladie. J'en viens à présent au deuxième enjeu de ce texte, la création d'une cinquième branche en faveur de la prise en charge de l'autonomie. En 2060, les personnes de plus de seront près de 5 millions, contre 1,4 million aujourd'hui. Le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie passera de 1,2 million en 2015 à 2,2 millions Quand on a de l'espoir, la vieillesse même est belle », écrivait Anton Tchekhov. Nous sommes confrontés à un formidable enjeu de société, celui d'accompagner au mieux nos aînés, de leur offrir une qualité de vie digne et épanouissante. Les sénateurs du groupe du RDSE plaident depuis de très nombreuses années pour la mise en place d'une grande réforme de la dépendance. Nous saluons donc cette mesure. Mais si l'on peut se réjouir que cette réforme soit enfin à l'ordre du jour, nous sommes plutôt réservés quant à la méthode choisie créer une cinquième branche par le biais d'un amendement dans un projet de loi sur la dette sociale semble pour le moins incongru. Pour mémoire, le système à quatre branches a été institutionnalisé il y a vingt-six ans par la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. La création d'une cinquième branche est donc une réforme de grande ampleur, qui aurait mérité de faire l'objet d'un projet de loi à part entière ou, tout du moins, d'être examinée dans le cadre du prochain projet d'autant que, comme l'a rappelé notre président Alain Milon, « son financement n'est pas assuré, ses bénéficiaires ne sont pas connus et sa gouvernance n'est pas définie S'agissant de son financement, justement, si je salue l'affectation de près de 2,4 milliards d'euros à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour amorcer le chantier, je crains que cette enveloppe ne soit tout d'abord insuffisante. Selon les estimations du rapport Libault, publié en mars 2019, les moyens supplémentaires nécessaires s'élèveront en effet à environ 6 milliards d'euros en 2024 et à plus de 10 milliards d'euros Nous craignons par ailleurs que ce financement n'intervienne trop tard, à l'instar de la CNSA, qui a émis des réserves sur l'échéance de 2024, la jugeant « incompatible avec l'urgence de la mise en oeuvre d'une grande loi C'est pourquoi un amendement du groupe du RDSE visait à dégager de nouvelles ressources dès 2021 ; malheureusement, celui-ci a été déclaré irrecevable. Quoi qu'il en soit, soyez assuré, monsieur le secrétaire d'État, que le groupe du RDSE, le moment venu, sera attentif aux modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle branche pour qu'elle puisse impulser une véritable politique de l'autonomie à la hauteur des enjeux.

deux textes ambitieux et nécessaires, alors que la crise sanitaire et économique que nous traversons jette une lumière crue, à peine atténuée par l'engagement sans faille du personnel soignant, sur les limites et les faiblesses de notre système de santé. Cette crise a balayé d'un revers de main l'espoir de voir se résorber, d'ici à quatre ans, une dette sociale composée des déficits cumulés des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et disparaître avec elle la caisse chargée de son amortissement, la Cades. Créée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 pour une durée initiale de treize ans, la Cades a vu son existence prolongée à plusieurs reprises au rythme des transferts et des reprises de dette. La dernière en date remonte à 2010 après que la crise financière de 2008 a incité le gouvernement d'alors à transférer 130 milliards d'euros de dettes supplémentaires et à retarder son extinction La pandémie de covid-19 et les mesures de confinement mises en oeuvre pour en limiter la progression ont provoqué à la fois un effondrement des recettes et une hausse des dépenses comme rarement- si ce n'est jamais -auparavant. Pour sécuriser durablement le paiement des pensions et des prestations, une reprise par la Cades de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'Acoss, qui n'a pas vocation à porter de tels déficits, est donc inévitable. L'article 1 du projet de loi ordinaire relatif à la dette sociale et à l'autonomie prévoyait ainsi un nouveau transfert de dette pour un total de 136 milliards d'euros

L'article 1 du projet de loi organique, quant à lui, prolonge jusqu'en 2033, c'est-à-dire pour neuf années supplémentaires, la durée de vie de la Cades, ainsi que la mobilisation de ses recettes, à savoir la CRDS, une fraction de la CSG et une contribution du Fonds de réserve pour les retraites. Les textes adoptés par l'Assemblée nationale ont été partiellement modifiés lors de leur passage en commission. Parce qu'elle estimait que la prise en charge d'une partie de la dette des hôpitaux par la Cades devait incomber à l'État, la commission des affaires sociales est revenue sur cette disposition. Le débat est évidemment légitime et méritait d'être posé. Il ne nous semble cependant pas incohérent qu'une partie de la dette des établissements de santé soit considérée comme une dette sociale, dès lors que ce sont les caisses primaires d'assurance maladie qui les financent en grande partie. Il serait faux par ailleurs de considérer que les investissements réalisés ne l'ont été que dans l'immobilier. Pendant des années, en effet, les établissements de santé ont été encouragés à emprunter auprès des banques pour financer leurs besoins en raison d'un Ondam contraint. En effectuant ce transfert de dette dès 2021, les établissements de santé retrouveraient de la visibilité et des marges de manoeuvre, ce qui leur fait actuellement défaut. Notre groupe, attaché à cette opération de bonne gestion financière, a déposé un amendement visant à réaffecter une partie de la dette des hôpitaux à la Cades. Nous aurons, mes chers collègues, l'occasion d'en débattre dans quelques instants. Ces deux projets de loi ouvrent en outre la porte à la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale- et d'un nouveau risque donc - consacrée à la prise en charge de l'autonomie. Cette réforme, attendue de longue date par les professionnels de santé, est une avancée sociale majeure qu'il nous faut saluer : elle offrira une ossature aux politiques existantes, favorisera la mise en oeuvre de nouvelles mesures et encouragera une approche plus préventive de l'autonomie. Dès 2024, date à laquelle s'achèvera l'amortissement de la dette reprise par la Cades en 2010, une fraction de la CSG sera réorientée vers la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, majorant ainsi son financement à hauteur de 2,3 milliards d'euros. Le secrétaire d'État, Adrien Taquet, l'a rappelé : en 2040, près de 15 % de la population, soit environ 10,5 millions de personnes, auront

que viendront compléter à l'automne la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et, dans le courant de l'année prochaine, un projet de loi consacré au grand âge et à l'autonomie que nous souhaitons ambitieux. Nous nous félicitons également de l'adoption en commission de notre amendement visant à intégrer les associations de personnes en situation de handicap au sein des concertations que mènera, dans le cadre de sa mission, M. Laurent Vachey. Cette réforme ne doit, en effet, et en aucun cas, omettre la question du handicap. cette mission feront l'objet d'un rapport, remis en septembre prochain au Parlement, sur les conditions de création d'un nouveau risque et d'une nouvelle branche de la sécurité sociale. Il précisera notamment les conditions de leur financement à court terme. Cette réforme, faut-il le rappeler, est scrutée avec attention dans des territoires d'outre-mer vieillissants. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la part des personnes âgées de plus a été multipliée par 1,5 entre 1999 et 2014 et devrait continuer à croître dans les années à venir. Selon l'Insee, cette part devrait ainsi doubler dans les Antilles d'ici à 2030, pour représenter près de 30 % de la population. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, parce qu'une meilleure prise en charge de l'autonomie ne saurait attendre, parce qu'il y voit une avancée sociale majeure, le groupe La République En Marche votera en faveur des projets de loi organique et ordinaire relatifs à la dette sociale et à l'autonomie, sous réserve évidemment

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, après les différents projets de loi sur l'état d'urgence sanitaire et et leur flot d'ordonnances, et alors que nous sortons tout juste d'un épisode particulièrement traumatisant pour nos concitoyennes et nos concitoyens, les deux projets de loi organique et ordinaire qui nous sont soumis vont ni plus ni moins que plomber pour des années notre système de protection sociale.

à la Cades et pas reprise par l'État ? Comment justifier que ces 136 milliards d'euros vont être, en réalité, supportés et financés par les contribuables à travers la CSG et la CRDS, dont on sait pertinemment que ce ne sont pas des impôts progressifs ? Le Gouvernement, face à une situation d'ampleur exceptionnelle, fait le choix de se défausser et de confier ce gouffre financier à un organisme social. C'est d'autant plus insupportable que ces 136 milliards d'euros sont dus en grande partie au confinement généralisé de la population pendant deux mois, ce qui ne relève absolument pas de la responsabilité de la Cades. Si la pandémie explique pour une part ce confinement, la décision prise s'explique, au fond, par la tension qui pesait sur notre système hospitalier et son incapacité à faire face à l'afflux des patients. réalité douloureuse est la résultante de choix politiques assumés par le Gouvernement et ceux qui l'ont précédé : 10 milliards d'euros de restrictions budgétaires draconiennes en sept ans, réalisées sur le dos des hôpitaux, des milliers de lits fermés, des suppressions d'emplois à tour de bras. Mais regardons de plus près comment se déclinent ces 136 milliards d'euros de dette : une partie, à savoir 13 milliards d'euros, provient de la dette hospitalière. Or, sur la quasi-totalité des travées de la Haute Assemblée, nous sommes d'accord : les dépenses d'investissement des hôpitaux relèvent de l'État, et non de la sécurité sociale. Certes, notre commission des affaires sociales a supprimé ce dispositif, mais permettez-moi de dénoncer à la fois les mensonges du Gouvernement et son tour de passe-passe. En novembre dernier, le Premier ministre, après plus de neuf mois de grève de l'ensemble des services d'urgence de France, avait annoncé la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux par l'État et non par la sécurité sociale, comme vous vous apprêtez à le faire. Si je résume : vous transférez aux hôpitaux la dette que vous étiez censé reprendre à ces mêmes hôpitaux Encore une fois, alors que la Cades est alimentée par la CRDS et la CSG, nous considérons que ce n'est pas à nos concitoyennes et nos concitoyens de payer la crise liée au covid-19 ni les dettes hospitalières fabriquées par les gouvernements successifs. D'autant que, comme on l'a rappelé, les conditions dans lesquelles la Cades peut emprunter sont bien moins favorables que celles de l'État. C'est donc un choix aberrant économiquement, sauf à justifier de futures restrictions budgétaires. Alors Alors que la crise sanitaire a démontré qu'il était plus que jamais indispensable de consolider notre système de protection sociale, vous lui imposez, une fois encore, une surcharge financière indue et mortifère. Pour faire passer ce mauvais coup, vous faites semblant de tirer des leçons de la crise vécue par les personnes en perte d'autonomie dans les Ehpad ou à domicile. Vous allez donc créer une cinquième branche de la sécurité sociale. Mais pour quoi faire, monsieur le secrétaire d'État ? La sécurité sociale a été créée en 1945 par Ambroise Croizat et Pierre Laroque c'est un système de protection sociale qui couvre toute une vie, de la naissance à la mort, avec tous ses aléas. De notre côté, nous considérons que la perte d'autonomie, que ce soient les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, est liée à l'état de santé et, donc, que les dépenses doivent relever d'une branche existante, celle de l'assurance maladie.

Nous nous opposons à cette fiscalisation et à cette privatisation de la sécurité sociale, tout comme nous nous opposons à la non-compensation par l'État des exonérations de cotisations. Pour rappel, vous avez voté 66 milliards d'euros d'allégements l'an dernier, soit la moitié pile de la dette que vous appelez « sociale Bien entendu, nous ne sommes pas pour le. À l'inverse de cette cinquième branche qui dénature notre modèle social, nous proposons, comme l'a expliqué ma collègue Cathy Apourceau-Poly, la création d'un grand service public national de la perte d'autonomie et de l'accompagnement, incluant les établissements médico-sociaux et les aides à domicile. Ce service public national aurait pour vocation de revaloriser tous ces métiers, dont chacun a enfin pris conscience de l'importance durant la pandémie. Tous ces salariés, majoritairement des femmes, d'ordinaire invisibilisés et maltraités par la société, ont fait tourner le pays en étant en première ligne pendant le confinement.

2,3 milliards d'euros à l'horizon de 2024 ? Permettez-moi de citer le rapport Libault, qui a notamment souligné combien les enjeux liés au grand âge étaient exponentiels et estimé à 10 milliards d'euros le besoin de ressources supplémentaires en 2030. Pour répondre à ces défis, la sécurité sociale a besoin de financements, de recettes nouvelles.

vous l'aurez compris : nous sommes profondément hostiles à la marchandisation des services à la personne et de notre système de protection sociale. Vous ne serez donc pas surpris si notre groupe vote contre ces deux projets de loi.

Il convient de sécuriser le fonctionnement de l'Acoss en transférant le montant de 136 milliards d'euros à la Cades. La commission des affaires sociales a souhaité soustraire de ce montant le tiers de la dette hospitalière, c'est-à-dire 13 milliards d'euros, considérant que ces dépenses relevaient de la responsabilité de l'État.

il s'agit de préparer l'avenir de la sécurité sociale à travers la création d'une cinquième branche consacrée à l'autonomie. Cette disposition est la première pierre que nous posons pour la prochaine réforme du grand âge, qui permettra à notre société de s'adapter au vieillissement

La mise en place d'un service départemental des aînés et des aidants, avec une déclinaison territoriale par canton, permettrait d'instaurer une équité et un guichet unique de coordination des intervenants à domicile auprès des personnes âgées dépendantes. Cela permettrait de renforcer la prévention, mais aussi de coordonner tous les intervenants à domicile et de prévoir les sorties d'hospitalisation en amont. Par ailleurs, il convient de veiller à l'amélioration des conditions de travail en établissement, en créant plus d'emplois et en valorisant les professions d'infirmier et d'aide-soignant. Cela passera par la revalorisation des salaires, comme le ministre de la santé l'envisage, à hauteur de 6 milliards d'euros, ainsi que par un grand plan national de formation. En effet, la VAE est insuffisamment connue et l'apprentissage peu développé. Nous allons gravement manquer d'infirmiers et d'aides-soignants.

débuter il y a de très nombreuses années. Je voudrais rappeler que Philippe Bas, ministre de la santé de Jacques Chirac en 2006, préconisait de parvenir à un taux d'encadrement d'un employé par pensionnaire en 2012. Enfin, la crise sanitaire a encore davantage mis en évidence la très grande fragilité et la précarité du secteur du maintien à domicile.

un mot particulier pour le rapporteur de la commission des affaires sociales, qui est un expert des questions de financement et qui est aussi toujours à la recherche d'une forme de sagesse et d'équilibre. Qu'il en soit remercié. Ma collègue Jocelyne Guidez abordera la question de l'autonomie. Pour ma part, je traiterai celle du financement de notre dette sociale, qui est une problématique majeure pour notre pays,

À sa création, en 1996, la Cades avait pour objectif de rembourser la dette accumulée par la sécurité sociale à l'échéance de 2009. Nos prédécesseurs avaient même créé un prélèvement dédié-

pour couper le robinet alimentant la dette sociale. La première orientation s'explique simplement : la dette hospitalière a servi à financer des investissements qui appartiennent à l'État. Or la Cades n'a pas été conçue pour cela, mais pour amortir les déficits de financement de la branche maladie.

ce que ne peut faire la Cades, et à meilleur taux. C'est à lui qu'il revient de prendre en charge la dette hospitalière et non à la Cades. Je soutiens pleinement l'amendement de notre rapporteur en ce sens. En ce qui concerne la règle d'or, les textes actuels prévoient que le législateur peut autoriser un régime à recourir à des ressources non permanentes, telles que l'emprunt, mais uniquement pour satisfaire des besoins de trésorerie et non pour couvrir des besoins de financement. Il faut appliquer ces dispositions

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il n'y a pas de cohésion nationale sans fraternité, ni de fraternité sans solidarité. Notre héritage républicain, fidèle à la pensée de Victor Hugo, nous exhorte à considérer que rien n'est solitaire, mais que tout est solidaire. Le lien intergénérationnel au coeur de nos discussions est le pivot de tout modèle social qui veut inscrire son action dans l'équité et la justice. Aussi, la dépendance et le soutien aux personnes âgées ou en situation de handicap constituent un enjeu vital. J'emploie volontairement le mot « enjeu », et non « problématique », car ces questions sont tout sauf une problématique. Elles sont partie intégrante de notre société. À l'aune du vieillissement de la population, notre réponse doit être ambitieuse. En somme, si la question de l'espérance de vie est importante, celle de l'espérance de vie en bonne santé l'est d'autant plus. Par ailleurs, répondre aux défis de la dépendance et de l'autonomie, c'est aussi se préoccuper de toute cette chaîne de personnes qui les accompagnent au quotidien. Les proches aidants constituent une pièce centrale du puzzle : ils doivent assumer à la fois des obligations professionnelles et d'autres, censées être plus « naturelles ». Ils doivent parfois faire face à de lourdes maladies comme Alzheimer. Surmenage, épuisement psychologique, manque de répit : les besoins sont immenses. Prenons garde, mes chers collègues, qu'ils ne redeviennent pas les grands oubliés. C'est également se soucier des professionnels, tout aussi indispensables, comme les auxiliaires de vie. Des mesures devront être prises tant sur l'attractivité de leur profession et sur la formation que sur la revalorisation des salaires.

Par ailleurs, cette mise en place n'entraîne aucune modification des modalités de financement de la prise en charge de la dépendance et aucune nouvelle ressource n'y est substantiellement affectée. La question de l'opportunité de ces deux textes se pose donc très clairement, en particulier du point de vue des bénéficiaires, lesquels, à ce stade, ne tireront aucun bénéfice de cette nouvelle Pour autant, au-delà du symbole, la création d'une cinquième branche sera l'occasion, pour le Gouvernement, de porter une politique financière dédiée au grand âge et à l'autonomie qui existera en tant que telle, sans être dépendante de l'évolution de l'Ondam. Mais encore faut-il des financements et une meilleure visibilité quant au calendrier. Or le transfert de 0,15 point de CSG entre la Cades et la CNSA ne satisfait pas les besoins financiers. Cette affectation permettrait de majorer les financements de la CNSA à hauteur de 2,3 milliards d'euros par an, mais pour quelles actions, sachant que le rapport Libault estimait le besoin à 10 milliards d'euros ? Enfin, ce transfert n'interviendra qu'en 2024. Pourquoi attendre trois ans ? Même si des concertations sur les conditions de financement à court terme devraient avoir lieu, on s'interroge sur ce qui pourra être mis en oeuvre prochainement et sur les moyens déployés. Sur ce point, ce texte n'apporte aucune réponse. Cette date permet tout simplement d'assurer le maintien de l'existence de la Cades. Ainsi, alors que notre pays a besoin de plus d'accompagnement, la prochaine loi de financement de la sécurité sociale offrira-t-elle des mesures suffisantes ?

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ces textes nous arrivent de l'Assemblée nationale avec rien de moins qu'une nouvelle branche de sécurité sociale, consacrée à l'autonomie. Il faut saluer une telle ambition dans le domaine médico-social, si souvent affichée depuis quinze ans et si rarement concrétisée. Elle porte la promesse d'une couverture du risque de perte d'autonomie plus large, plus cohérente, plus juste, financée de manière plus pérenne. Cette promesse peut-elle être tenue ? Il faut d'abord s'interroger sur la capacité à faire de ceux qui la portent. À cet égard, la méthode qui nous est proposée n'est pas rassurante. Le texte initial contenait un ensemble de dispositions déjà peu faites pour conjurer le scepticisme : un rapport à la rentrée sur la faisabilité du chantier du cinquième risque, une nouvelle annexe aux et un financement devant être pris, dans quatre ans, dans les comptes déjà négatifs de la Cades. Tel était le projet du Gouvernement sur l'autonomie, dans un texte consacré d'abord au remboursement de la dette sociale La nouvelle annexe aux lois de financement de la sécurité sociale s'impose : nous ne votons pour l'heure en loi de financement de la sécurité sociale que sur une vingtaine de milliards d'euros de crédits, alors que la dispersion des financeurs porte le montant global des dispositifs existants à près de 66 milliards d'euros. Nous avons donc incontestablement besoin d'une vision des choses un peu plus large. À l'Assemblée nationale, nos collègues députés ont créé, sans concertation préalable, un cinquième risque et une cinquième branche de la sécurité sociale, et ils ont confié immédiatement sa gestion à la CNSA. C'est à l'évidence prématuré, puisque le rapport censé éclairer la décision ne sera rendu qu'en septembre. Les députés ont d'ailleurs avancé sa date de publication. publication. Comment rédiger un rapport complet sur ce sujet, en si peu de temps, durant l'été, sans oublier la concertation nécessaire avec tous les acteurs de ce secteur ? Je crains que le rapport ne soit incomplet, notamment sur la question des financements. Mais admettons que l'on encadre le tableau avant de l'avoir peint. Admettons que l'on crée le cadre de gestion avant de savoir ce que l'on financera et comment on le financera. Le plus dur reste à faire : rendre plus efficace notre système d'intervention et lui donner les moyens de fonctionner. Il faudra pour cela répondre à un certain nombre d'interrogations. La nouvelle branche, intitulée « autonomie », a donc vocation à regrouper les prestations et services destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. D'après D'après APF France handicap, 35 millions de personnes pourraient à terme être concernées : 12 millions de personnes en situation de handicap, 15 millions de personnes âgées et 8 millions de proches aidants. C'est un défi considérable qu'il nous faut collectivement relever. Sur la prise en charge du grand âge, tout a été dit ces dernières années. Las, l'épidémie de covid-19 a donné un écho fantastique au silence avec lequel ont été accueillies- pour l'instant -les propositions des rapports Libault, El Khomri ou celles de nos collègues Bonne et Meunier au nom de notre commission des affaires sociales. Les chantiers sont nombreux : il faudra augmenter le taux d'encadrement des personnes accueillies en établissement, hisser les professionnels du secteur au moins au niveau du SMIC, investir massivement, améliorer la coordination des acteurs, construire une politique de prévention plus efficace ... J'en oublie Le monde du handicap s'interroge également sur les opportunités qu'ouvrirait une telle innovation. Au premier abord, harmoniser les dispositifs d'aide à l'autonomie permettrait d'exaucer enfin le voeu émis par le législateur en 2005, qui prévoyait la suppression de toutes les barrières d'âge dans un délai de cinq ans. Plus de quinze années ont passé, et il est, par exemple, toujours impossible de faire une demande de PCH si le handicap est survenu après 60 ans, puisque l'on est alors réputé éligible aux prestations destinées aux personnes âgées. L'extension annoncée de la prestation suscite par ailleurs de grands espoirs qu'il pourra être opportun de concrétiser dans ce nouveau domaine de la sécurité sociale. Sur le périmètre et le calcul des prestations, mais aussi sur le reste à charge zéro, sur l'accès aux droits et aux aides techniques, sur la simplification des aides à l'aménagement du logement ou au transport, et pour ne rien dire de la gouvernance du secteur du handicap, les marges de progression sont encore nombreuses. Sur tous ces points, notre commission a fait des propositions. L'inclusion de cette politique dans le périmètre de la sécurité sociale offre d'intéressantes perspectives. Reste à les concrétiser. De plus, en décloisonnant les dispositifs destinés aux personnes âgées et handicapées, une politique unifiée de l'aide à l'autonomie permettrait d'améliorer la couverture des besoins, de compenser plus adéquatement les pertes d'autonomie, bref de rendre plus universel le soutien de la Nation aux plus vulnérables. sur tout cela, il nous faudrait des garanties. D'abord, sur le partage des tâches : le rôle des départements dans la politique médico-sociale est quasiment séculaire et n'est contesté par personne. Le dialogue qu'ils entretiennent avec l'État, notamment les ARS, devra être clarifié. Le rôle des aidants, qui accomplissent un travail informel d'une valeur presque égale aux crédits médico-sociaux votés en PLFSS, devra également être pris en compte. Notre commission a d'ailleurs précisé que le rapport attendu pour septembre devra être précédé d'une consultation de tous les acteurs du médico-social, dont les collectivités locales et les aidants. Il faudra enfin des garanties sur le financement de cette nouvelle branche, qui nécessitera des ressources cinq fois plus importantes que celles prévues à l'article 2. Là encore, notre commission a fait des propositions qui méritent l'intérêt. Nous serons au rendez-vous des prochaines discussions budgétaires. À défaut de telles clarifications, les frustrations seront immenses, et cette création apparaîtra pour ce qu'elle est : une promesse de plus. Nous serons vigilants sur l'issue de ces travaux. Le Sénat est prêt à être un acteur bienveillant

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon collègue Yves Daudigny a exprimé, en début de discussion générale, la ferme opposition de notre groupe à ces projets de loi. Pour ma part, j'évoquerai les questions relatives à la perte d'autonomie. Ce n'est une surprise pour personne, il existe bien un besoin social concernant la prise en charge de la dépendance liée à l'âge. Le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie a déjà été évoqué : il traduit la longévité de notre population, ce dont il faut se réjouir. Mais nous savons que cette ultime période de la vie peut être source d'inquiétude, pour les plus vieux comme pour leurs proches et leur famille. La survenue des premiers signes de perte d'autonomie frappe la population de façon inégale, à des âges plus ou moins avancés. La prise en charge financière est complexe : l'évaluation du degré de dépendance est fixée par les grilles GIR- les groupes iso-ressources. Elles ne sont, il faut en convenir, qu'un instrument administratif d'affectation du soutien de la compensation que peuvent fournir les secteurs sanitaire et médico-social, l'aide apportée par les auxiliaires pour les gestes du quotidien au domicile et, pour les aînés les plus dépendants, dans les Ehpad. Le reste à charge des coûts pour les bénéficiaires est varié. Il dépend du degré de dépendance, des ressources personnelles et du lieu de prise en charge. Par ailleurs, le vieillissement est une source de fatigue pour les aidants, le conjoint ou les enfants, qui s'usent prématurément, « par porosité », comme le souligne la philosophe Cynthia Fleury. Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire d'un : la reconnaissance d'une cinquième branche et du risque « autonomie » doit permettre une meilleure couverture des frais nécessaires et une sanctuarisation des moyens. Il existe un risque de perte d'autonomie lié à l'âge : ne plus pouvoir s'habiller seul, découper sa viande, laver son assiette, remplir son caddie Décrite ainsi, il est évident que la perte d'autonomie peut survenir à tout âge de la vie, dès lors qu'on est affecté par un handicap. Pour les socialistes, le risque « autonomie » doit intégrer cette dimension. C'est l'occasion de lisser les différences de droit selon que l'on entre ou pas dans l'une ou l'autre des cases. Ce risque lié au handicap est à ce jour insuffisamment couvert. C'est ce que nous dit le collectif Handicaps, lequel formule des recommandations auxquelles il faudra répondre : droit universel dès la petite enfance, reste à charge zéro, financement assuré par la solidarité nationale, équité sur les territoires, respect des droits et choix des individus concernés ... Le secteur associatif devra être associé aux futurs travaux Mes chers collègues, l'adaptation de la société au vieillissement n'est pas un enjeu nouveau et n'a pas été laissée de côté par les précédents gouvernements : c'était d'ailleurs l'intitulé de la loi que nous avons portée. Elle a permis de changer de regard sur cette tranche d'âge, a impulsé une dynamique de prévention et de lutte contre l'isolement. La loi a également relevé les plafonds de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile pour près de 700 000 bénéficiaires. Résolus à poursuivre dans cette voie, les socialistes sont favorables, pour la gestion de ce nouveau risque, à la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale. Le premier enjeu sera d'assurer une gestion démocratique, paritaire, plaçant les usagers au coeur des décisions. Le second enjeu est évident : il s'agira d'assurer des recettes suffisantes à cette nouvelle branche.

D'autres pistes devront être évoquées : financement par la branche maladie, avec d'autres cotisations ; de la solidarité nationale ? Il faut le dire, monsieur le secrétaire d'État, nous sommes dans le flou face à cette improvisation soudaine du Gouvernement. Vous profitez d'un transfert de dette sociale inacceptable pour poser la première pierre d'un chantier pharaonique. Nous ne sommes pas dupes de vos intentions. Nous craignons que vous ne bâtissiez que le rez-de-chaussée d'une branche de la sécurité sociale et qu'il revienne aux futurs assurés sociaux d'étayer le financement par des complémentaires « autonomie », sources d'injustice sociale et de creusement d'inégalités. Pour toutes ces raisons, si la maîtrise d'ouvrage vous revient, sachez que la maîtrise d'oeuvre devra compter sur toutes les énergies vigilantes, dont la nôtre. La parole est à M.

madame Meunier,

Une telle décision hypothéquerait l'avenir de nos assurances sociales, en leur faisant supporter inutilement et injustement la « dette covid », dont elles ne sont pourtant pas responsables, alors que cette dette pourrait être plus habilement gérée par l'État.

L'accès universel aux soins, la garantie de prestations sociales permettant de maintenir le niveau de vie et l'assurance d'un revenu de remplacement en cas de perte d'emploi sont autant d'atouts qu'il nous faut renforcer et élargir. la crise sanitaire a également révélé des fragilités, qui sont le fruit d'un sous-financement chronique organisé depuis de longues années, en particulier de nos hôpitaux et de nos Ehpad, en première ligne face à l'épidémie. L'article 1 du projet de loi organique prévoit le organique prévoit le report de la fin du remboursement de la dette sociale prévue en 2033 et, en même temps, le transfert de 136 milliards d'euros de dette à la Cades.

après la crise de 2008, avait transféré 130 milliards d'euros de dette à la sécurité sociale. Sous couvert d'impératif budgétaire pour préserver les finances sociales, cette opération permettra demain au Gouvernement de maintenir sous pression pour de longues années les dépenses de santé. En effet, ce sont 17 milliards d'euros de CRDS et CSG qui auraient pu servir à financer des politiques sociales, au moment où nos concitoyennes et concitoyens en ont le plus besoin. Cette dette est d'autant plus injuste qu'elle sera remboursée uniquement par les salariés, les demandeurs d'emploi et les retraités. Les entreprises, en revanche, ne participeront pas à l'effort collectif. Pourtant, qui a profité de l'activité partielle et des garanties de l'État ? Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 1 du

Je n'entrerai pas dans une longue explication, car celle-ci a déjà été donnée. Le report de la date limite d'amortissement de la dette est nécessaire pour permettre de nouveaux transferts, sans alourdir sensiblement les prélèvements obligatoires. Quel

fondamental de notre système de sécurité sociale, puisqu'il assure la pérennité de son financement. C'est aussi la contrepartie logique de l'autonomie financière de la sécurité sociale : la dette sociale doit être gérée par la sécurité sociale et non pas transférée à l'État,

la réalité. La situation actuelle est exceptionnelle par la soudaineté et l'ampleur de cette crise. Toutefois, comme en 2011, le déficit sans précédent de la sécurité sociale qui s'annonce pour 2020 résultera principalement, vous le savez, d'une contraction de l'assiette de ses recettes.

à un nouveau transfert de dette vers la Cades, dont les conditions de financement sont proches de celles de l'État, je l'ai dit précédemment. Transférer cette dette à l'État remettrait en cause le principe vertueux du remboursement de la dette et reviendrait à considérer que l'État doit assurer le financement de la sécurité sociale. Surtout, cela reviendrait à changer les règles du jeu, alors même que nous ne sommes pas encore sortis de la crise et que l'instabilité économique est bien réelle. Enfin, tout en s'engageant à rembourser la dette, le Gouvernement choisit aussi de financer des priorités

qui veut que les déficits sociaux soient transférés à une caisse qui en assure l'amortissement avec des recettes sociales.

en ces circonstances exceptionnelles, n'est-il pas autorisé de s'interroger ? Vous-même, monsieur le rapporteur, écrivez dans votre rapport, à la page 68 : « En soi, une durée de vie de la Cades, désormais fixée à

présenter l'amendement n° 4. Le fait de soumettre la sécurité sociale aux règles de discipline budgétaire imposées par le pacte de stabilité dans la zone euro est évidemment un vieux fantasme des libéraux. Il semble que ce fantasme prenne corps aujourd'hui, par le biais de l'article 1 introduit par la droite sénatoriale en commission des affaires sociales. Sous couvert de bonne gestion de la sécurité sociale, il s'agit d'interdire tout transfert de dettes complémentaires à la Cades. Désormais, non seulement on ferme le robinet à l'arrivée, en plaçant l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'Ondam, sous le niveau des dépenses, mais aussi on met un couvercle sur la sécurité sociale.

comment voulez-vous que la sécurité sociale puisse continuer à fonctionner normalement ? Les parlementaires qui voteront cet article seront tenus pour responsables, je l'ai déjà dit, des fermetures de lits, des fermetures de services et de la dégradation des soins dans leurs territoires. La droite sénatoriale ne semble pas avoir tiré les enseignements de la pandémie de covid-19, qui peut revenir

vous le savez très bien, pour qu'une règle soit crédible, surtout en matière financière, il faut qu'elle soit stable. Si l'on commence à la remettre en cause le lendemain du jour où on l'a votée,

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

Cet article vise à modifier le cadre organique des lois de financement de la sécurité sociale en matière d'information du Parlement et de mesures relatives à la dette.

Si la volonté première de la majorité sénatoriale est de circonscrire cette dette à une dette patrimoniale- elle serait constituée en grande partie par des investissements immobiliers -, il faut le dire, ces investissements ne sont pas uniquement immobiliers ; durant des années, les établissements de santé ont été encouragés à emprunter auprès des banques pour financer leurs besoins. Le

Aussi, ce transfert intervenant dès 2021, les établissements de santé retrouveront rapidement des marges de manoeuvre indispensables pour réinvestir au bénéfice de la santé de nos concitoyens. Il est donc de bon sens, nous semble-t-il, de réintégrer cette reprise de dette des établissements de santé. Cet amendement vise, à cet cet effet, à rétablir deux alinéas portant sur une clarification de la nature des dispositions facultatives des lois de financement de la sécurité sociale relatives à la dette sociale, en indiquant que ces dispositions doivent doivent avoir un effet sur la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et sur son amortissement. Nous restons ainsi dans la cohérence des positions que j'ai développées par ailleurs.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

projet de loi organique prévoit qu'une nouvelle annexe au PLFSS permettra d'intégrer au texte la présentation des dépenses relatives à l'aide à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. La commission des affaires sociales de votre assemblée a adopté un amendement visant à compléter ces dispositions organiques pour que l'annexe fasse figurer les dépenses relatives à la prévention, à l'apprentissage de l'autonomie et à la recherche. Il s'agit évidemment d'enjeux majeurs- nous ne pouvons que vous rejoindre sur ce point -, qui pourront être abordés en tant que de besoin dans cette nouvelle annexe, dont le contenu pourra évoluer. Mais, d'une part, ces enjeux

Le scrutin est clos.

Gréaume, sur l'article. L'article 1 prévoit un transfert de dette d'un montant global de 136 milliards d'euros à la Cades. Je pense, mes chers collègues, qu'il est temps que le Gouvernement explique aux Français ce qu'est véritablement la dette sociale.

Rétablir clairement la distinction entre la dette sociale et la dette de l'État empêchera ce mécanisme de culpabilisation, avec un « trou de la sécu » qu'il faudrait absolument combler, et ce au prix d'une perte de droits pour les assurés sociaux et d'un affaiblissement de la sécurité sociale. En transférant ce montant à la Cades, ce sont près de 18 Il est trop facile d'inclure dans la dette sociale des charges qui devraient être assumées par l'État et de s'en servir ensuite comme justificatif afin de réduire les dépenses

plus de 130 milliards d'euros de dette à la Cades. Nous pensons que ce transfert met en danger la sécurité sociale pour les années à venir

qui est ici remise en cause. En effet, les travaux immobiliers et les investissements de rénovation afférents ont jusqu'à présent toujours relevé du budget de l'État. Soit le Gouvernement décide aujourd'hui de transférer cette dette à la sécurité sociale, mais, dans ce cas, il transfère les compétences et surtout les dotations correspondantes soit le Gouvernement ne transfère pas ces compétences, mais, dans ce cas, il assume le remboursement de la dette liée aux investissements. Vous ne pouvez pas décider de faire payer à la sécurité sociale les

celle des retraites par points par exemple, ainsi que les fermetures d'hôpitaux, les fermetures de services et la diminution des prestations sociales. Alors que s'achève bientôt le Ségur de la santé, j'espère, monsieur le secrétaire d'État, que vous avez eu le courage de dire aux représentants des professionnels de santé que leurs conditions de travail vont encore se dégrader dans les prochaines années en raison de cette dette à rembourser. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 1. Quel

1,2 milliard d'euros proviennent du déficit cumulé de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui régit notamment le régime spécial des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. le Gouvernement pour financer ce déficit est donc de le faire reprendre par la Cades. Mais si le déficit de la CNRACL a été aggravé, c'est bien parce que les gouvernements successifs ont décidé de geler le point d'indice des fonctionnaires et de ne pas remplacer les départs à la retraite.

prélevés sur les salaires et 22 milliards d'euros sur les pensions de retraite, les 10 milliards d'euros restants provenant essentiellement des placements financiers et des prélèvements sur le patrimoine. On voit donc bien l'injustice du recours à la CSG, qui revient à faire financer la future branche perte d'autonomie

payer. De l'argent, il y en a : il suffit de se donner les moyens d'aller le chercher ! Par cet amendement, nous réclamons donc la création, en lieu et place de la CASA, d'une contribution

collectif et solidaire. Nous avons déjà rappelé les enjeux de la perte d'autonomie pour aujourd'hui et pour les années à venir. Pour y faire face, nous pensons qu'il est indispensable de disposer d'un service public et d'un financement public pour assurer une couverture intégrale de la perte d'autonomie. À défaut, les familles continueront à acquitter de lourds restes à charge et les assureurs privés pourront s'enrichir au détriment des assurés sociaux.

considérant que confier la gestion de ce nouveau risque à une branche de la sécurité sociale « impliquerait l'effacement du département et le transfert de la gestion des prestations à un des réseaux existants de caisses locales De même, dans le projet de loi initial relatif à la dette sociale et l'autonomie, il n'était question que d'un rapport sur la pertinence de la création d'une cinquième branche associée au cinquième risque. Or nous voici en présence de quatre alinéas qui créent directement cette cinquième branche telle démarche est contraire aux principes mêmes de la sécurité sociale. Je passe sur le fait que la perte d'autonomie serait plutôt le neuvième risque ... En effet, elle relève, selon nous, de la branche maladie. Les séparer, c'est créer une nouvelle strate fragilisant l'ensemble, avec des transferts de crédits, et tourner le dos à l'expertise

Enfin, sortir la perte d'autonomie et la dépendance de la branche maladie conduit à substituer de nouveaux prélèvements fiscaux aux cotisations sociales assises sur la richesse créée par le travail. Comme pour la CSG, la fiscalisation casse la dynamique de solidarité intergénérationnelle, ce qui isole les différents bénéficiaires des aides de la société. Au-delà des slogans, il y a des réalités. La prise en charge de la perte d'autonomie mérite

une réforme en profondeur de la prise en charge de perte d'autonomie. Il a, d'une part, procédé à une réaffectation d'une fraction de CSG à la CNSA, et, d'autre part, proposé la remise d'un rapport sur les conditions de création d'un nouveau risque ou d'une nouvelle branche de sécurité sociale relative à l'aide à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Les députés ont souhaité aller plus loin que le projet initial du Gouvernement, en élargissant dès à présent le champ des risques couverts par la sécurité sociale à la perte d'autonomie et en créant une cinquième branche de sécurité sociale.

et un solde financier, de mettre en évidence l'effort national qui y est consacré et de garantir un équilibre. Au-delà du pilotage financier, c'est aussi et surtout le moyen de mieux définir les règles de pilotage et de gestion propres à ce risque. C'est donc une étape indispensable pour assurer un réel pilotage et une bonne couverture de ce risque social, ce qui est précisément l'objectif du Gouvernement pour garantir une meilleure prise en compte de la perte d'autonomie. Rien n'est préempté quant au financement et à la gouvernance de cette nouvelle branche. La concertation sur le pilotage et la

Nous devons être à la hauteur de l'enjeu. Nos aînés, nos concitoyens en situation de handicap et les aidants nous regardent. La création d'une nouvelle branche peut être décidée dès aujourd'hui : « chiche », suis-je tenté de dire.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Cette nouvelle branche doit permettre la mise en place d'une véritable politique d'accompagnement des personnes en situation de dépendance, afin qu'elles puissent conserver leur autonomie le plus longtemps possible. Cela doit notamment passer par une réforme de la tarification des établissements médico-sociaux, tout particulièrement des Ehpad. En effet, si l'espérance de vie augmente, le gain se réduit souvent, malheureusement, à des mois passés en mauvaise santé. De plus en plus de personnes âgées se retrouvent en situation de perte d'autonomie à leur domicile, parce qu'elles n'ont pas les moyens de financer leur hébergement en établissement. Il est donc nécessaire de résoudre la question du reste à charge, beaucoup trop lourd pour de nombreuses familles. Dans cette perspective, nous proposons que le rapport que le Gouvernement remettra le 15 septembre prochain examine les conditions d'une réforme de la tarification des établissements médico-sociaux, en vue de la réduction de ce reste à charge.

un très grand nombre de questions relevant de la politique de prise en charge de la perte d'autonomie, dont celle de la tarification des établissements sociaux. La création d'une nouvelle branche et d'un nouveau risque relatifs à la prise en charge de la perte d'autonomie s'accompagnera de différentes réformes de fond,

L'urgence est à la relance de notre pays par le renforcement des services publics, mais vous préférez poursuivre dans la voie des exonérations de cotisations sociales, qui ont fait perdre 90 milliards d'euros à la

complètement vide, financée par les assurés sociaux eux-mêmes. Bref, comme l'a dit notre collègue Pierre Dharréville à l'Assemblée nationale, il s'agit d'une « belle opération publicitaire, loin de l'histoire de la sécurité sociale

sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux est parvenue à l'adoption d'un texte commun.